tendant à créer une commission d'enquête afin d'évaluer l'intervention des services de l'État dans la gestion des conséquences environnementales, sanitaires et économiques de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, de recueillir des éléments d'information sur les conditions dans lesquelles les services de l'État contrôlent l'application des règles applicables aux installations classées et prennent en charge les accidents qui y surviennent ainsi que leurs conséquences et afin de tirer les enseignements sur la prévention des risques technologiques, présentée

L'État se doit d'être transparent. L'information dont il dispose- pour autant qu'elle soit connue et fiable -doit être clairement et précisément délivrée à nos concitoyens, aujourd'hui submergés par des torrents de fausses informations qui alimentent un climat de méfiance. La réponse du Parlement se doit d'être à la hauteur de l'enjeu majeur que constitue la protection de l'environnement et des populations, en particulier lorsqu'il s'agit de la gestion des accidents industriels. En matière de prévention, cet accident soulève la question des évolutions récentes du droit de l'environnement, qui, sous couvert de simplification, paraissent aboutir à une régression au coup par coup des exigences imposées aux activités industrielles potentiellement dangereuses. Je pense notamment au passage de nombreuses ICPE du régime de l'autorisation à celui de l'enregistrement ou de la déclaration, à la sortie d'un grand nombre de projets de l'évaluation environnementale, alors même que la France fait l'objet d'une mise en demeure de la Commission européenne, à la remise la remise en cause de l'indépendance de l'autorité environnementale et à la faiblesse du montant des sanctions prononcées en matière de droit pénal de l'environnement. L'ensemble de ces choix politiques doit nous alerter, car simplifier ne peut en aucun cas aboutir à remettre en cause la sécurité des activités ayant un impact sur l'environnement. En l'occurrence, nous avons appris que l'extension des capacités de stockage de produits dangereux a été autorisée sans évaluation environnementale. Pourquoi ? De même, l'État ne disposait pas d'une connaissance exacte des substances dangereuses présentes sur le site. Pourquoi ? Cette commission d'enquête devra impérativement répondre à ces questions et à beaucoup d'autres afin d'apporter des solutions concrètes. La réglementation environnementale n'est pas une variable d'ajustement économique, avec plus de 1 000 sites Seveso dans notre pays. Toutes les leçons de cet événement devront être tirées. C'est la raison pour laquelle le groupe du RDSE soutiendra, bien évidemment, la création de cette commission d'enquête.

Celle-ci est indispensable pour comprendre les failles qui ont conduit à cet accident industriel majeur, ainsi que les dysfonctionnements dans la gestion de la crise qui n'est pas encore derrière nous : des éleveurs, des agriculteurs font face à l'interdiction de commercialisation de leur production, touchée par les suies. C'est une bataille de tous les instants que nous menons à leurs côtés pour faire en sorte, par exemple, que le lait soit collecté ou que leurs pertes soient indemnisées, ce qui n'est toujours pas le cas. Gestion de crise qu'il faut concevoir dans la durée avec l'évaluation des risques, le suivi épidémiologique au long court, l'état des sols et de l'eau à long terme. Nous nous réjouissons que nos demandes répétées conduisent à l'installation, demain, en Seine-Maritime, d'un comité de suivi regroupant les différents acteurs, y compris les citoyens. Par la voix de la présidente de notre groupe, nous en avons appelé à la transparence, dans cet hémicycle, dès le lendemain de l'incendie, dans l'indifférence totale- -de la ministre présente. Nous avons ensuite assisté à des déclarations différentes, voire divergentes de membres du Gouvernement, rendant inaudible, voire suspecte, la parole de l'État et traduisant un recul inacceptable de ce dernier face aux enjeux. Nous souhaitons que cette commission d'enquête fasse toute la lumière sur les premiers instants- déterminants -de la gestion de la crise. Pourquoi les sirènes ont-elles retenti plusieurs heures après le début de l'incendie ? Pourquoi les élus locaux ont-ils été mis sur la touche, alors qu'ils sont les premiers relais d'information auprès des populations ? ? À nos yeux, la commission d'enquête devra aussi se fixer d'autres objectifs, et pas des moindres : comprendre pourquoi ce drame est survenu, en évaluant notamment les conséquences du détricotage du droit de l'environnement et de la sûreté

enfin améliorer encore les plans de prévention des risques technologiques en donnant à l'ensemble des acteurs- représentants des salariés, élus locaux, services de l'État -les outils nécessaires pour prévenir ce type d'accident et protéger les

-et de nombreuses communes du Pays de Bray, du nord de la Seine-Maritime et, plus largement, des départements voisins ont vu s'élever dans le ciel un nuage noir, épais, nauséabond à la suite de l'incendie de l'usine Lubrizol, classée Seveso seuil haut nous l'avons appris depuis, de l'entreprise voisine, Normandie Logistique, consommant plus de 9 000 tonnes de produits hydrocarbures et de produits divers. Les retombées du nuage ont tapissé de particules et de suie les jardins, les cours d'école, les récoltes des agriculteurs- les empêchant de vendre leurs produits -, les bâtiments et les véhicules. Les fumées ont indisposé nombre d'habitants, encore inquiets pour leur santé. Les communications des services de l'État, distillées au fil de la journée, se sont voulues rassurantes, mais les élus et la population sont restés légitimement inquiets. Il s'est écoulé de nombreuses heures entre le déclenchement du feu et l'activation des sirènes d'alerte. Des maires disent ne pas avoir été informés. Les consignes de confinement ont été confuses. Les informations sur la dangerosité potentielle du sinistre ont tardé La population a eu le sentiment que quelque chose lui était caché, ce qui a suscité défiance et colère. L'enquête judiciaire déterminera- au plus vite, je l'espère -l'origine, les causes de l'incendie et les responsabilités des uns et des autres. La commission d'enquête parlementaire que nous appelons de nos voeux

Cette commission d'enquête devra également déterminer si l'intervention des services de l'État a été conforme aux dispositions réglementaires et s'il n'était pas possible de mieux et plus rapidement informer les maires et la population. Comme en 2011 après AZF, cette commission d'enquête doit permettre un retour d'expérience, proposer, le cas échéant, des pistes d'amélioration du contrôle des installations industrielles à risque, des processus d'alerte des autorités locales et de la population et mesurer la quantité et la qualité des moyens engagés pour évaluer les conséquences environnementales et sanitaires d'un tel sinistre. Pour toutes ces raisons, et pour concourir à la plus totale transparence, cette demande de commission d'enquête nous paraît non seulement recevable, mais indispensable. Nous voterons, bien évidemment, cette proposition

Elle vise, d'une part, à évaluer l'intervention des services de l'État dans la gestion de la crise, dans ses conséquences environnementales, sanitaires et économiques et, d'autre part, à recueillir des informations quant aux conditions dans lesquelles ces mêmes services ont contrôlé les règles applicables aux installations classées dans quelle mesure ils prennent en charge les éventuels accidents. Nous comptons, comme cela a été souligné, 1 312 installations classées Seveso en France, réparties dans un grand nombre de départements.

Gironde est le département qui compte le plus de sites sensibles. Il s'agira, plus globalement, de tirer les enseignements sur la prévention des risques technologiques et d'évaluer les dispositifs d'alerte qui encadrent les sites industriels Seveso.

associera toutes les parties prenantes- collectivités, professionnels, agriculteurs, associations de protection de l'environnement, riverains, professionnels de santé, parlementaires ... -dans le suivi des conséquences à court et moyen terme. Il est fondamental d'informer, et ce de la façon la plus transparente possible, les personnes touchées et de répondre aux inquiétudes des citoyens et des élus locaux, qui peuvent légitimement s'interroger sur les risques et les mesures de sécurité appliquées afin d'éviter qu'une telle crise ne se reproduise.

pour explication de vote. Le 26 septembre dernier, les habitants de la métropole rouennaise se réveillaient dans un immense nuage de fumée noire provenant de l'incendie de l'usine Lubrizol, classée Seveso seuil haut. Poussé par des vents dominants, le panache de fumée, long de vingt kilomètres, se déplaçait rapidement vers l'est et touchait plus de 200 communes, dont 112 en Seine-Maritime.

L'intervention rapide et le très grand professionnalisme des secours ont permis de maîtriser le sinistre dans la matinée et d'éviter les victimes, malgré des risques majeurs. Le plan particulier de prévention, déclenché rapidement par la préfecture de Seine-Maritime, a permis d'adopter un certain nombre de mesures de sécurisation et de mesures sanitaires d'urgence. alors que la Seine-Maritime est le département qui compte le plus de sites Seveso- près de quarante -après les Bouches-du-Rhône, la culture du risque reste insuffisante : nombre d'habitants ne savaient pas à quoi correspondaient les sirènes actionnées à huit favorisé une anxiété collective que les premiers messages, qui se voulaient rassurants, des services de l'État n'ont pas permis d'atténuer. Les informations nombreuses, mais peu coordonnées et parfois contradictoires, malgré la volonté forte de transparence du Gouvernement, n'ont pas réussi à rassurer les populations, d'autant moins que cette chaîne d'information a oublié un maillon fort : les maires, prévenus tardivement et souvent de manière très imprécise. Quinze jours plus tard, de nombreuses questions restent en suspens. Une telle catastrophe aurait-elle pu être évitée ? Comment agir face à un tel accident industriel ? Quelles sont et quelles seront les conséquences sanitaires, environnementales, économiques et agricoles réelles ? La commission d'enquête demandée par le président Retailleau et soutenue par l'ensemble des présidents de groupe et des présidents de commission doit permettre de faire toute la lumière sur l'intervention des services de l'État dans la gestion des conséquences environnementales, sanitaires et économiques de l'incendie de l'usine Lubrizol et d'en tirer toutes les conséquences pour développer une véritable culture du risque majeur. Elle doit également permettre d'évaluer les modalités d'application des directives Seveso et d'en tirer, surtout pour l'avenir, tous les enseignements utiles. Le groupe Les Républicains votera, bien évidemment, cette proposition de résolution. La parole est à M. Claude Malhuret, pour explication de vote. Les causes de l'incendie de l'usine Lubrizol, le 26 septembre dernier, ne sont pas encore connues. Elles font l'objet d'une enquête de police judiciaire qui a débuté mardi dernier. Je voudrais d'abord rendre hommage au travail remarquable des pompiers et des services de secours qui sont intervenus dans des circonstances très difficiles et qui sont parvenus rapidement à éteindre cet incendie. certainement permis de limiter l'ampleur de cet événement. Aurait-on pu faire mieux ? C'est tout l'objet de la commission d'enquête que nous souhaitons unanimement créer. Il faut en effet que nous tirions toutes les leçons de cet accident pour pouvoir en empêcher d'autres. Pour cela, il nous faut évaluer l'action des services de l'État avant, pendant

concerne la gestion de l'incendie, nous savons déjà que l'information des maires et des habitants peut sans doute être améliorée. Nous essaierons de savoir comment. En aval ensuite, nous nous interrogerons sur la gestion des conséquences de l'accident. Nous savons qu'elles sont multiples : environnement, santé et économie. Là encore, l'information est un sujet majeur. Nos concitoyens demandent légitimement la plus grande transparence sur le résultat des analyses en cours, comme le Gouvernement s'y est engagé. Le groupe Les Indépendants votera cette proposition de résolution afin que le Sénat puisse contribuer à la recherche de pistes d'amélioration pour qu'un tel événement ne se reproduise pas.

parole est à M. Éric Gold. Si les conseils communautaires comportent encore trop peu de femmes en leur sein, la situation est encore moins satisfaisante dans les exécutifs de ces conseils. Ainsi, seulement 8 % de femmes président une intercommunalité et 20 % sont présentes dans les exécutifs intercommunautaires.

Ainsi, d'une part, dans le cas d'un nombre impair de membres du bureau, la différence entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes ne devra pas être supérieure à 1 ; d'autre part, s'il n'est pas possible pour des raisons numériques de respecter cette règle, il faudra que chaque sexe soit représenté proportionnellement à son nombre dans le conseil communautaire. Cet amendement permettra ainsi de féminiser la tête des intercommunalités et d'avancer de façon réaliste. Merci dès lors que l'élection des membres par fléchage permet une composition paritaire de l'organe délibérant. La France a été le premier pays à adopter une loi fondée sur l'application du principe paritaire pour les élections. Il s'agit de la loi du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. Grâce à l'adoption de contraintes légales, la parité progresse au sein de la majeure partie des assemblées locales et de leurs bureaux, à l'exception notable des intercommunalités, qui ne sont concernées par aucun dispositif contraignant. D'après les données 2017 du ministère de l'intérieur, seulement 34 % des élus communautaires sont de sexe féminin. Par ailleurs, 20 % des postes de vice-président sont attribués à des femmes et 8 % sont présidentes d'exécutif.

cet amendement a pour objet de favoriser la parité au sein des bureaux des conseils communautaires, dans la limite des possibilités numériques.

place. Ce n'est pas à vous que je dois le rappeler, l'égalité entre les hommes et les femmes est l'une des grandes causes du quinquennat. Si vous me permettez ce mauvais jeu de mots, pour vous comme pour la majorité de cette assemblée et pour les rapporteurs, c'est un petit peu « la parité si je mens En effet, alors que, au titre de l'article 1 de notre Constitution, « la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électifs et aux fonctions électives », ce texte ne comporte aucune mesure prévoyant de telles dispositions.

les obligations que l'on doit respecter pour constituer le bureau de l'intercommunalité, puisque celle-ci est un espace de consensus et de projets partagés, notamment sur la gouvernance.

dont le nombre est égal à 20 % du nombre de conseillers communautaires, la parité, en permettant que les vice-présidents soient élus en prenant

très peu représentées : 8 % en sont présidentes et 20 % sont présentes dans les exécutifs. Même lorsque la parité est assurée dans les assemblées délibérantes, elle l'est rarement dans les organes exécutifs. Elle est délicate à atteindre dans les EPCI, nous l'avons vu, mais cela ne doit pas être une raison de diminuer encore davantage la part de femmes dans le bureau exécutif. Aussi, par cet amendement de bon sens, nous proposons que la proportion de femmes au sein des exécutifs soit au moins équivalente à leur proportion au sein de l'organe délibérant. Cela permettra de renforcer la représentativité des femmes et leur prise en compte dans les instances de décisions, notamment dans les exécutifs. Cela permettra aussi de diversifier leurs champs d'action,

n'est pas incompatible, tant s'en faut, avec ce que nous avons défendu précédemment. Car si le nombre de femmes membres de l'exécutif intercommunal

-qui nous permettra vraisemblablement d'adopter dans quelques instants notre amendement et celui de la commission. Je souligne simplement, pour rétablir les faits,

menées notamment par les gouvernements précédents, avec les lois de 2013 et de 2014 sur la parité. Malheureusement, comme l'a dit ma collègue Annie Guillemot, seuls 16 % des maires sont des femmes, seulement 30 % d'entre elles siègent au sein des EPCI et moins de 9 % sont présidentes d'une intercommunalité. La parité en politique consiste surtout, pour les hommes, à céder la place aux femmes. ils ne le font que lorsque la loi les y oblige. Là où il y a une contrainte légale, les femmes représentent à peu près la moitié des élus. Mais là où il n'y a pas de contrainte légale, tel n'est malheureusement pas le cas. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement,

sur la question de la place des femmes dans les intercommunalités aujourd'hui, c'est l'impossibilité de conclure de vrais accords locaux, ce qui entraîne, de fait, une disproportion entre

à ses certitudes et libre de voter comme il l'entend. Je ne crois pas que l'on pourra trouver une solution pour la cause des femmes. À tout le moins, on pourra en trouver une pour la parité, mais pas forcément pour les dames.

34 % de femmes dans les conseils communautaires, 20 % seulement dans les exécutifs et 92 % d'hommes présidents d'EPCI. On pourrait penser que les choses progressent.

une alternance systématique dans les fonctions exécutives entre le premier vice-président et le président de façon à obtenir systématiquement une représentation paritaire à la tête de l'exécutif

depuis le début du mois de janvier à la création de la communauté et au changement de président- trois mois plus tard -, pour simplement élire les membres de cette institution ! J'appelle votre attention sur les dommages

des territoires et dans l'organisation de chaque intercommunalité.

D'autres choses sont à faire. Monsieur le ministre, vous avez accepté par anticipation de réfléchir à l'idée de la représentation par liste dans les communes de moins de 1 000 habitants. C'est un élément qu'il faudra mettre en place rapidement.

on peut imaginer qu'il est possible d'élire l'ensemble des membres du bureau, après le président et les vice-présidents, de manière simplifiée.

Si le nombre de candidatures déposées correspond exactement au nombre de postes à pourvoir, les candidats sont immédiatement élus, comme c'est actuellement le cas pour la commission permanente des conseils départementaux. Sinon, la règle actuelle s'appliquerait.

Aujourd'hui, ils sont élus au scrutin secret uninominal à la majorité absolue, comme le prévoit la circulaire du 13 mars 2014 relative à l'élection et mandats des assemblées et des exécutifs municipaux Cependant, nous avons tous observé sur le terrain que le régime actuel de cette élection pouvait être considérablement chronophage. Il représente généralement plusieurs dizaines de votes et s'avère particulièrement lourd à mettre en oeuvre lors des conseils d'installation pour un enjeu souvent minime.

selon les configurations locales, leur nombre est important et leur élection particulièrement fastidieuse, alors même que très souvent un consensus politique a été trouvé en amont par les élus et qu'il n'y a qu'un candidat par poste. Le présent amendement vise donc à ce qu'un appel à candidatures soit ouvert sur l'ensemble des postes des autres membres du bureau, en dehors du président et des vice-présidents. Si le nombre de candidatures déposées correspond exactement au nombre de postes à pourvoir, les candidats sont immédiatement élus, comme c'est actuellement le cas pour la commission permanente des conseils départementaux.

et le scrutin de liste à la proportionnelle nous paraît peu compatible avec l'esprit de consensus qui doit présider à la nomination des membres du bureau, autres que le président et les vice-présidents. Nous avons longuement débattu de ce sujet

Pour les communes de moins de 1 000 habitants soumises au scrutin majoritaire, il existe une contrainte exigeant que les conseillers communautaires soient le maire, les adjoints, puis les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. Or cette exigence n'a pas de réelle justification. En effet, il n'existe aucun lien entre la composition d'un exécutif municipal et les compétences de l'intercommunalité. Selon quels principes un maire devrait-il définir l'ordre de ses adjoints et leurs compétences en fonction de l'intercommunalité ? Par ailleurs, les communes de moins de 1 000 habitants disposent rarement d'un nombre important de sièges à l'intercommunalité. L'argument selon lequel l'ordre du tableau fait apparaître les conseillers les mieux élus en premier après le maire, les adjoints et les conseillers municipaux délégués ne peut donc pas tenir lieu de justification. Pour une plus grande souplesse, il est proposé de reconduire les anciennes modalités en laissant au conseil municipal le soin de désigner les conseillers communautaires lors de son installation et ainsi de les modifier au cours du mandat si besoin est. Cette rédaction permettrait de résoudre l'objectif de l'article, à savoir garantir la présence des maires dans les conseils des EPCI. Quel

dès le premier mandat ou après deux ou trois mandats, des responsabilités, y compris dans l'exécutif de l'intercommunalité. L'idée, c'est de détendre un peu le dispositif pour permettre un choix

part proportionnelle, on peut aboutir à une situation dans laquelle un conseiller communautaire était plus bas sur la liste par rapport à son rang que sur le volet de la liste des conseillers municipaux. Je ne sais pas si je suis clair en disant

la mission de l'élu local ne conserve son sens et sa richesse qu'à la condition qu'il l'exerce au niveau communal et au niveau intercommunal. Le projet de loi prévoit de renforcer le rôle du maire au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

que l'administration territoriale de proximité repose désormais sur le couple complémentaire communes-intercommunalité. Il est indispensable de consacrer dans la loi- il serait même préférable que ce le soit dans la Constitution -la complémentarité entre commune et intercommunalité au sein du groupe communal ou groupe local.

il est proposé de consacrer de façon indéfectible la complémentarité au sein du groupe communal, en prévoyant que les élus communautaires émaneront toujours des communes. émaneront toujours des communes. Cette question est essentielle : le changement de mode de scrutin qui couperait le lien entre communes et intercommunalité transformerait les maires en chiens de garde, sans moyens, puisque l'essentiel de ce qui concerne leur territoire se passerait ailleurs et sans eux.

du CGCT, pour l'enrichir et préciser le lien de complémentarité du couple communes-intercommunalité, ce qui est fondamental. Ainsi, le premier alinéa de cet article pourrait être rédigé ainsi Les métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes, qui constituent avec leurs communes membres un groupe local par leurs liens de complémentarité et d'interdépendance,

C'est exactement l'intention de la commission des lois, qui se traduit dans des actes, par tout ce que nous faisons depuis que nous sommes ici, et dans les propositions à venir.

qui est plus

Or, en cas d'extension du périmètre communautaire ou de fusion en cours de mandat, le nombre de sièges d'une commune peut être réduit à un. Si cette commune compte 1 000 habitants ou plus, le conseil municipal élit alors le nouveau conseiller communautaire, ainsi que son suppléant à partir de listes devant comporter deux noms. Mais si le suppléant élu à cette occasion démissionne ensuite de son mandat de conseiller municipal, le conseil municipal ne peut pas élire un nouveau suppléant. Cet amendement tend à remédier à cette situation. La

un suppléant au conseil communautaire dans les communes qui ne disposent que d'un siège. Lorsqu'il y a lieu en cours de mandat de procéder à une nouvelle répartition des sièges au sein de l'organe délibérant de l'EPCI- nous avons évoqué cette question pour les communes concernées -, chaque commune doit alors réélire ses représentants. Les communes de plus de 1 000 habitants le font parmi les membres du conseil municipal qui ont été fléchés. Les communes qui ne disposent que d'un seul siège élisent également un suppléant, sur le modèle de ce qui est fait, comme cela a été rappelé, lors de la désignation des conseillers communautaires communautaires à l'occasion du renouvellement général. Les amendements prévoient que, si le mandat de ce suppléant cesse, le conseil municipal élit un nouveau suppléant. La loi pourvoit déjà au cas où il n'y a plus de suivant de liste pour remplacer un conseiller communautaire. Lorsque la commune ne dispose que d'un siège et s'il n'y a plus de suppléant, le conseiller communautaire est remplacé par le premier conseiller municipal élu sur la liste correspondante au conseil municipal et qui ne figurait pas sur la liste des candidats au conseil communautaire. Toutefois, la commission des lois admet qu'il pourrait être opportun de permettre au conseil municipal, dans le cas très limité qui fait l'objet des amendements, de choisir son futur conseiller communautaire. Mais il nous paraît, à ce stade, difficile de trancher le sujet

pour respecter ce principe. Cet amendement vise donc à combler un « trou dans la raquette », celui d'un ancien maire resté conseiller municipal et conseiller communautaire. Dans cette configuration, l'ancien maire toujours membre du conseil municipal est chargé de représenter sa commune au conseil communautaire. Or s'il vient à démissionner de son mandat de conseiller communautaire, celui qui sera désigné à sa place est non pas le premier dans l'ordre du tableau, mais celui qui suit le démissionnaire. Cette Cette situation absurde revient à exclure des maires ou des adjoints du rôle de conseiller communautaire qui devrait leur revenir. Il est donc proposé d'y remédier de manière très simple en supprimant du code électoral la mention « qui le suit », afin que soit bien désigné le premier dans l'ordre du tableau qui n'est pas déjà conseiller communautaire.

en cours de mandat, même s'il était conseiller communautaire et que la loi actuelle lui permet de ne plus être maire mais de rester conseiller communautaire, sera imposée une réélection

est à M. Jean-Pierre Grand, sur l'article. Je tenais à me féliciter de l'adoption de nouveau par le Sénat de mon amendement permettant de mettre fin à l'incompatibilité entre le mandat de conseiller communautaire et l'exercice d'un emploi salarié au sein d'une commune membre.

Cela ne concerne en rien le mandat de conseiller municipal : un salarié d'un EPCI ou d'une commune peut se porter candidat et exercer un mandat municipal au sein d'une autre commune, membre du même EPCI. Il aura toutefois à choisir entre son emploi en tant qu'agent de l'EPCI et l'exercice de ce mandat, s'il est également élu conseiller communautaire. Il devra, afin de faire cesser l'incompatibilité, démissionner de son poste de salarié communal ou démissionner de son mandat de conseiller communautaire. Les mandats de conseiller municipal et de conseiller communautaire diffèrent. En toute logique, les régimes d'inéligibilités et d'incompatibilités ne peuvent être confondus. C'est pourquoi le RDSE s'oppose à l'élargissement de ce dispositif aux salariés d'EPCI

supprimer l'incompatibilité entre le mandat d'élu communautaire et l'exercice d'un emploi de salarié de l'EPCI ou des communes membres ? Cela me paraît très compliqué. Je préférerais, comme le président Requier, qu'on s'en tienne au texte actuel.

avec l'exercice de tout emploi salarié au sein non seulement de l'EPCI, mais également dans l'une des communes membres. À l'inverse, rien n'empêche un conseiller municipal de travailler au sein de l'EPCI. Il existe donc une sorte d'inégalité d'inégalité de traitement. Le ministère de l'intérieur a répondu à une question écrite sur ce sujet : il a reconnu la dissymétrie ou l'asymétrie de traitement entre le conseiller municipal et le conseiller communautaire

J'essaie d'imaginer la situation dans laquelle un agent territorial d'une commune est élu conseiller municipal et communautaire dans une autre commune, membre de la même intercommunalité et peut donc devenir le collègue de son patron. Pourquoi pas ? Il peut même exercer une fonction dans l'exécutif communautaire, voire la fonction suprême de président de cette intercommunalité, tout en étant l'agent territorial d'un maire membre de cet EPCI. Je ne fais aucun procès d'intention, et après tout, je le redis, pourquoi pas ? Néanmoins, il est bon d'avoir des règles claires. Pour éviter toute forme de difficultés particulières, il existe ces règles d'incompatibilité. Nous ne les introduisons pas dans le droit à l'occasion de ce projet de loi.

pour considérer que l'objet de ce texte est de replacer le maire au coeur de l'intercommunalité. Je vais vous donner un exemple : un agent territorial est élu dans une autre commune, dont il devient le maire. Il est aujourd'hui confronté à l'interdiction de siéger comme conseiller communautaire : on empêche un maire du territoire intercommunal d'être conseiller communautaire, alors que l'interaction entre la commune qu'il représente et l'intercommunalité est reconnue par toutes et tous. C'est la raison pour laquelle il faut lever cette incompatibilité et permettre à des employés d'une commune, par ailleurs élus dans une autre, de siéger à l'intercommunalité, s'ils sont maires.

Merci